Monsieur le président,

nous ne pouvons pas continuer nos travaux sans faire écho à la colère populaire qui s'exprime. Certains se plaisent à ne commenter que les actes de violence. Nous condamnons toutes et tous, et avec force, ces violences sans précédent et nous avons toutes et tous été choqués par des images montrant des individus, souvent des « ultras », s'attaquant à des symboles de l'histoire de notre pays, mais ces violences ne sauraient faire oublier le message clair que des milliers de nos concitoyennes et de nos concitoyens envoient au Président de la République

Mes chers collègues, le peuple de France en colère ne demande ni la lune ni des miettes, il réclame la justice sociale, maintenant, pas dans trois mois Satisfaire pour le moins ces deux revendications, c'est possible, et c'est possible maintenant ! Ici, au Sénat, ne nous faisons pas complices des choix du Président de la République et de son gouvernement. Oh ! Nous sommes des parlementaires, nous sommes la représentation nationale, dont se méfient aujourd'hui nos concitoyennes et nos concitoyens, qui placent maintenant les enjeux démocratiques au coeur de leurs revendications. Envoyons un signal à celles et ceux qui souffrent dans notre pays ! Chers collègues, la France traverse une crise sociale et institutionnelle et nous en sommes à à voter des mesures dont l'impact va aggraver la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Ils n'en veulent pas ! Refusons de continuer à débattre d'un budget qui n'apporte aucune réponse concrète à la colère citoyenne, mais qui, à l'inverse, va accroître les souffrances humaines. Ce matin, je vous demande, monsieur le président, de réunir une conférence des présidents. Face à la gravité de la situation, et alors que le Premier ministre va recevoir les partis politiques et leurs représentants au Parlement, nous devons exiger de sa part des engagements concrets. C'est une C'est une nécessité ! Aujourd'hui, pour être à la hauteur de sa sagesse, le Sénat devrait porter la voix du peuple

les crédits de la mission « Outre-mer » que nous examinons ce matin présentent une double diversité : la diversité des collectivités auxquelles ils sont destinés, d'abord, puisqu'ils concernent au total onze territoires,

En 2019, cette stabilité se confirme, car, même si le montant total des crédits connaît une forte hausse, de plus de 20 % en crédits de paiement et de plus de 22 % en autorisations d'engagement, cette augmentation exceptionnelle est en réalité issue de deux importantes mesures

Il est cependant important de rappeler que les crédits de la mission « Outre-mer » ne représentent pas la totalité de l'intervention de l'État. Ces crédits comptent en effet pour moins de 15 % de l'ensemble des crédits budgétaires transversaux,

tel que retracé par le document de politique transversale, est donc en augmentation de plus de 4 % en autorisations d'engagement par rapport à 2018, et de plus de 1,5 % à périmètre constant. Comme chaque année, l'examen des crédits de la mission met en évidence des points positifs, mais aussi des motifs d'inquiétude. L'importante mesure de périmètre que j'ai évoquée a pour objet de permettre au Gouvernement

avons effectué en 2016 un contrôle budgétaire de ce dispositif de financement des investissements publics dont nous avons noté, avec tous les acteurs locaux, la souplesse de mobilisation et la capacité à initier rapidement des projets jugés essentiels

Une évaluation objective et partagée des dépenses fiscales ou sociales avant leur mutation en crédits budgétaires est toujours nécessaire, compte tenu de l'impact important que pourraient avoir des baisses de ressources sur la situation de l'emploi, dans un contexte de chômage de masse touchant plus particulièrement la jeunesse de chacun de nos territoires. Moins d'une année après la publication du Livre bleu outre-mer et après l'adoption, en 2017, de la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, il était nécessaire de mettre en place les premiers financements destinés aux contrats de convergence et de transformation qui découlent de ces deux dispositifs complémentaires. Ces financements au titre de la politique contractuelle de l'État totalisent pour 2019 un montant additionnel de 23 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 15 millions d'euros en crédits de paiement. Ils devront impérativement faire l'objet d'une montée en charge durant les prochains exercices afin d'atteindre les objectifs ambitieux assignés à la mise en oeuvre de ces deux textes. Considérant que ces plans se substitueront aux contrats en cours, qu'il s'agisse des contrats de plan, des contrats de développement ou des contrats de projets, avec un périmètre budgétaire élargi, il conviendra d'être particulièrement vigilant sur le respect des engagements financiers de l'État en fin d'exécution des conventions.

S'agissant des autres domaines d'intervention- logement, action sociale et sanitaire, action de formation, notamment au travers du service militaire adapté -, le temps qui m'est imparti ne permet pas d'entrer dans une analyse détaillée. J'indiquerai succinctement que l'on peut relever dans l'ensemble un maintien des moyens budgétaires alloués. Le budget qui nous est présenté pour 2019 se caractérise, en réalité, par sa stabilité ; il progresse même légèrement, contrairement à certains de ceux qui ont été votés durant la précédente décennie. On peut s'en réjouir, au moins s'en satisfaire, dans un contexte de contrainte budgétaire, en notant que ces crédits représentent pour 2019 0,54 % du budget de l'État, contre 0,48 % en 2018.

s'agissant du rattrapage des écarts de développement avec la métropole, nécessitent un effort financier nettement plus important de l'État, qui ne s'est pas totalement concrétisé pour 2019. Je rappelle que, pour certaines collectivités, cet écart, calculé en points de PIB par habitant, représente un retard de plus de 60 par rapport à la métropole, avec des taux de chômage compris entre 25 % et 30 %, voire plus de 50 % pour les jeunes, et une part de la population éligible au logement social atteignant parfois près de 80 %. En définitive, ce budget préserve les grands équilibres dans le financement des principales interventions de l'État en outre-mer, dans une optique de continuité. Il suscite, ne le nions pas, des inquiétudes, notamment en ce qui concerne les opérations de périmètre, lesquelles sont toujours sensibles, s'agissant de la transformation de dépenses fiscales ou sociales en crédits budgétaires et de la nécessaire validation concertée des volumes de ressources financières à transformer. Il porte les premiers crédits destinés à financer les actions résultant de la mise en oeuvre des dispositions de la loi de programmation relative même si l'on peut regretter leur insuffisance, au regard des enjeux de rattrapage économique et social dont tous les parlementaires ont souligné la gravité. Pour toutes ces raisons, et tout en étant, comme vous, conscient de l'importance des efforts qui restent à fournir pour permettre aux outre-mer de réduire les écarts de développement qui se sont creusés avec la métropole, je vous propose d'adopter les crédits de la mission « Outre-mer ». La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues rapporteurs, mes chers collègues,

À périmètre constant, le budget de la mission pour 2019 respecte donc la programmation pluriannuelle. Celle-ci aurait dû, au contraire, être réévaluée après la tenue des Assises des outre-mer, lesquelles ont permis de définir la stratégie ultramarine du quinquennat et le niveau réel des besoins de la mission « Outre-mer Le maintien de cette trajectoire est regrettable, d'autant qu'il entre en contradiction avec l'objectif de rattrapage des territoires ultramarins, fil conducteur du Livre bleu outre-mer. Certes, les crédits de la mission « Outre-mer » connaissent une hausse sensible-

correspondent à un transfert au profit du programme 138, « Emploi outre-mer », lié à la mise en oeuvre des exonérations de charges spécifiques. Il s'agit de mesures très décriées, vraiment loin de faire l'unanimité, qu'il nous faut donc accueillir avec une certaine prudence. La suppression de la TVA NPR et l'abaissement du plafond de réduction d'impôt sur le revenu devraient représenter des gains budgétaires atteignant respectivement 100 millions d'euros et 70 Le Gouvernement prévoit de mobiliser l'équivalent de cette dépense fiscale en dépense budgétaire afin de favoriser le développement économique des territoires et d'abonder le FEI. Cette logique est Cette logique est toutefois à double tranchant, puisque, si le caractère pilotable des dépenses budgétaires permet un meilleur ciblage que la dépense fiscale, il n'offre toutefois aucune garantie ni quant à leur réaffectation totale ni quant à leur pérennité.

Aussi, je souhaite que ces engagements soient, cette fois, spécialement surveillés, notamment par un contrôle budgétaire, afin de veiller à leur bonne exécution.

Après d'âpres échanges ici même, le projet initial du ministère des outre-mer a été corrigé sur certains points afin d'éviter que cette réforme ne se traduise par une trappe à bas salaire.

Les espoirs des entreprises guyanaises se portent désormais, madame la ministre, sur votre promesse d'examen au cas par cas, qu'il vous faudra tenir. Mon dernier point portera sur la somme de 1,7 milliard d'euros non ventilée dans le document de politique transversale. De quoi s'agit-il ? Comment et quand sera-t-elle affectée ? des contrats de convergence, qui doivent entrer en application en janvier 2019 ? Madame la ministre, il faut faire vite, car nos territoires en ont grandement besoin.

veux pouvoir compter sur vous. Je voterai donc les crédits de cette mission, mais une extrême vigilance s'imposera

La situation est particulièrement alarmante en matière de logement : au fil des ans, les crédits sont stables ou affichés en hausse, mais la construction ralentit pour un certain nombre de raisons, parmi lesquelles la complexité du parcours administratif figure en bonne place. Notre premier message, qui vaut aussi pour la défiscalisation, porte sur la nécessité de fluidifier les procédures pour favoriser le climat de confiance avec les opérateurs et leur permettre de consacrer plus de temps à leur coeur de métier. Ensuite, le Gouvernement propose, pour 2019, de greffer sur cette reconduction deux recyclages, lesquels ont suscité des réactions inédites par leur nombre et leur intensité. J'ai écouté les acteurs ultramarins pour analyser l'impact économique réel de l'ensemble de la tuyauterie sociale, budgétaire et fiscale pour 2019 et suggérer des réajustements. Le premier recyclage a surpris les Ultramarins. Au sortir des Assises des outre-mer et après la publication du Livre bleu outre-mer, l'État nous propose en effet une démarche budgétaire de recentralisation.

comptable, les chiffres sont à peu près équivalents, mais, économiquement, les subventions sont lentes à se mettre en place et les crédits sont volatiles d'année en année, alors que les suppressions de compensations fiscales sont pérennes

D'une part, on se demande encore s'il ne manque pas quelque 180 millions d'euros, peut-être parce que les calculs du Gouvernement se sont fondés non pas sur le CICE exigible, mais sur le CICE constaté, ce qui revient à pénaliser de fait certaines entreprises ultramarines qui n'ont pas exercé leur droit. D'autre part, D'autre part, la concentration au voisinage du SMIC va certainement « booster » l'embauche dans un premier temps, mais risque, à l'avenir, d'enfermer les outre-mer dans la « smicardisation » et les productions de moyenne gamme, alors qu'il faut aussi aider les entreprises à retenir les talents ultramarins pour mener l'offensive sur les activités à haute valeur ajoutée. Le Sénat a cependant voté des mesures de rééquilibrage en matière de réduction du coût du travail ainsi que des réaménagements fiscaux. Sous réserve de leur prise en compte, il nous est apparu logique de ne pas nous opposer à l'adoption des crédits de la mission « Outre-mer » pour 2019.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la plupart des outre-mer, face à une situation sociale très dégradée, constituent de véritables poudrières. Nous le vérifions en ce moment même : La Réunion s'est embrasée devant des mesures qui risquent d'accroître encore la cherté de la vie. Ces événements font suite aux émeutes survenues en Guyane, aux manifestations contre l'insécurité à Mayotte, aux urgences sécuritaires et sanitaires à Saint-Martin. Comment pourrait-il en être autrement, alors que le chômage des jeunes concerne plus de la moitié d'une génération, alors que plus de 110 000 logements sont insalubres dans les départements et régions d'outre-mer, alors que la mortalité infantile à Mayotte et en Guyane atteint un niveau Dans ces conditions, il ne suffit pas de se déplacer sur le terrain ou d'organiser de nouvelles assises. Madame la ministre, vous avez, certes, écouté les attentes immenses des outre-mer ; encore faut-il que les actions mises en oeuvre traduisent une réelle prise de conscience. Or nous craignons que la plupart des mesures annoncées en ce début de quinquennat ne restent à l'état programmatique. Les Assises des outre-mer se sont tenues huit ans après les états généraux de 2009, alors que les propositions formulées à l'époque n'ont rien perdu de leur actualité.

Notre commission s'est employée à rechercher la traduction de ces annonces dans le budget proposé. Dans le champ social, le bilan est bien mince : les crédits dédiés au logement et à la formation sont toujours en stagnation, de même que la maigre ligne budgétaire consacrée au sanitaire et au social.

Notre commission n'est pas opposée par principe aux mesures de périmètre touchant la mission. La conversion de mesures fiscales en crédits budgétaires peut être positive, à condition de réaliser au préalable la prédominance de la dépense fiscale n'est pas un choix des outre-mer, les budgets ayant été historiquement construits de cette façon. Prenons donc garde à ne pas asphyxier les économies ultramarines par un sevrage trop brutal. Votre rapporteur est cependant opposée à la mesure touchant à l'impôt sur le revenu. Mal évaluée, celle-ci ne pourra répondre au problème des inégalités, qui résultent avant tout de la cherté de la vie. Si la commission des affaires sociales n'a pas émis un avis défavorable sur ces crédits, c'est uniquement parce que, en réalité, ce budget ne comprend pas grand-chose à quoi nous pourrions nous opposer, dans la mesure où l'architecture budgétaire conduit la plupart des mesures touchant aux outre-mer à être opérées en dehors de cette mission.

Une discussion a également eu lieu sur les exonérations de charges, Georges Patient l'a évoquée et je ne vais pas insister. Une solution de compromis a été trouvée,

la suroccupation des établissements, l'absence d'activités proposées, l'isolement des détenus et l'accès difficile aux soins ont pour conséquence une grande violence, tant entre détenus qu'à l'égard des personnels pénitentiaires. Au vu de ces difficultés, il me semble indispensable de mettre en oeuvre une politique ambitieuse, avec trois objectifs principaux. Le premier est de mieux prendre en compte les spécificités des territoires ultramarins, notamment en transformant la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer en direction interrégionale, à l'image du dispositif en vigueur sur le territoire métropolitain, avec des moyens humains et financiers renforcés. Le deuxième objectif est de réduire la surpopulation carcérale. À cette fin, il me semble nécessaire de prévoir la construction de nouvelles places de prison, d'améliorer les alternatives à l'incarcération et de développer les conventions internationales bilatérales. Le troisième objectif est de favoriser la réinsertion des détenus. Cela implique un renforcement des moyens des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans nos territoires. Enfin, il importe de nouer un dialogue avec nos compatriotes ultramarins et de faire oeuvre de pédagogie pour faciliter une meilleure acceptation de la prison et lutter contre la fameuse loi d'airain dénoncée par notre ancien collègue Robert Badinter : en raison de leurs conditions de vie souvent difficiles, nombre d'entre eux

que le leur. Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention générale et le temps de l'explication de vote.

Elle vient aussi de l'attitude de l'État devant son obligation d'organiser la solidarité nationale. En effet, au lieu de s'appuyer sur la solidarité nationale, le Gouvernement ne fait que transférer les contributions des Ultramarins vers leur propre territoire. Toutes les mesures que nous avons combattues, comme la suppression de la TVA non perçue récupérable pour les entreprises et le resserrement de l'abattement sur l'impôt sur le revenu, seront,, financées par les Ultramarins eux-mêmes. Or nos territoires ultramarins souffrent d'un chômage chronique, structurel, important, insupportable. Madame la ministre, vous étiez voilà quelques jours à l'île de la Réunion, où plus de six jeunes sur dix sont au chômage vous avez pu constater la souffrance et le désarroi de la population réunionnaise, dont près de 42 % vit sous le seuil de pauvreté. Je vous félicite pour votre courage et pour l'écoute dont vous avez fait preuve vis-à-vis des Réunionnaises et des Réunionnais. Mais, vous l'aurez compris, il faut à présent aller vite, et beaucoup plus loin. Il faut que ces revendications soient entendues au plus haut niveau de l'État à l'image de cette crise sociale sans précédent qui secoue La Réunion, force est de constater que nos territoires d'outre-mer vivent actuellement dans la plus grande inquiétude. Cette situation doit s'améliorer rapidement, car les collectivités territoriales ne peuvent plus agir, en raison, notamment, de la contraction de la dotation globale de fonctionnement et de la suppression des contrats aidés. L'emploi en outre-mer devrait être la première priorité de cette mission ! Le programme 138 est, en ce sens, crucial. Pour l'essentiel, il prend en charge les exonérations de cotisations de sécurité sociale.

Sur le régime des aides directes aux entreprises de la nouvelle action n° 04, je m'interroge : pourquoi remplacer un dispositif qui fonctionne de façon relativement simple- la TVA non perçue récupérable -par une multitude de petits dispositifs complexes de soutien aux entreprises ?

J'en viens maintenant à nos compatriotes d'outre-mer, aux ménages touchés par la ponction de 70 millions d'euros par an prévue à l'article 4 du A-t-on évalué les effets de cette mesure sur la classe moyenne ? A-t-on pris en compte que ralentir un peu plus la consommation en outre-mer nous amènera tout droit vers de nouvelles crises sociales ? Le pouvoir d'achat, vous le savez, est l'une des principales préoccupations en outre-mer. L'État doit s'impliquer pour réduire les inégalités avec la métropole. Plusieurs propositions vous ont été faites, madame la ministre, parmi lesquelles la mise en place d'une continuité territoriale des biens et des marchandises, la révision de certaines taxes et le plafonnement des prix. Le débat doit être ouvert. Je pense que vous avez pleinement conscience des attentes de nos populations. Madame la ministre, nos outre-mer doivent surmonter à la fois l'éloignement géographique, l'insularité, l'étroitesse des marchés et l'exposition aux risques naturels.

n'est pas encore à la hauteur des enjeux de nos territoires ultramarins. En conséquence, nous nous abstiendrons sur les crédits de la mission.

pauvreté et précarité records, problèmes d'éducation alarmants, criminalité grandissante, manque d'infrastructures scolaires et hospitalières de quoi parle-t-on, mes chers collègues ? De nos banlieues ? De nos milieux ruraux ? D'un énième espace où l'État est en recul dans la France métropolitaine d'Emmanuel Macron ? Tout simplement d'autres territoires oubliés de la République, qu'on occulte bien trop souvent : les outre-mer. À l'appui du constat des grandes difficultés que ces régions des droits de l'homme sur l'effectivité des droits de l'homme dans les outre-mer fait état de situations d'extrême pauvreté auxquelles doit faire face une proportion élevée des populations ultramarines. L'exclusion sociale est provoquée notamment par un système éducatif limité, dont les répercussions ne peuvent être que négatives sur l'insertion socioprofessionnelle et le développement des territoires. Les infrastructures scolaires délabrées et mal réparties ne permettent pas aux jeunes d'avoir accès à une éducation de qualité. Sur le volet sanitaire également, le constat est préoccupant. Ainsi, le taux de la mortalité infantile et maternelle est largement supérieur à celui de la métropole. Pourtant, cette situation est décrite comme évitable, car la surmortalité serait due au manque de moyens dans les établissements hospitaliers et de mesures thérapeutiques. En outre, les spécificités climatologiques de ces territoires entraîneraient une prévalence des maladies infectieuses et parasitaires, couplées à un déficit d'accès à l'eau potable, notamment à Mayotte et en Guyane. Les enjeux de santé publique les plus élémentaires sont négligés, au détriment d'une population particulièrement exposée. Les régions et départements d'outre-mer ayant souffert trop longtemps du manque d'investissements de l'État et du recul des services publics, nous attendions beaucoup, madame la ministre, du budget qui leur serait alloué.

Dans ce budget, madame la ministre, vous faites le choix de doter massivement l'investissement privé pour l'emploi et les entreprises, au au détriment du programme « Conditions de vie outre-mer », au sein duquel nous constatons une réduction des financements accordés aux services publics et une stagnation de ceux alloués aux collectivités territoriales. Une fois de plus, vous appliquez votre, qui laisse entendre que le progrès social passe avant tout par une bonne santé économique, alors même que la pauvreté et la précarité de ces territoires exigeraient que l'on investisse davantage dans les services publics.

destiné à lutter contre les changements climatiques et à investir dans les énergies renouvelables. S'agit-il d'un acte manqué ? Au regard du climat majoritairement tropical des outre-mer et compte tenu du fait que la France est la deuxième puissance maritime mondiale, nous avions les moyens de devenir de devenir les champions des énergies propres, notamment hydraulique et solaire. Mais, une fois de plus, le Gouvernement est absent là où il aurait pu impulser une politique économique novatrice dans ces territoires. Mes chers collègues, par les résultats du référendum du 4 novembre dernier en Nouvelle-Calédonie, des Ultramarins ont renouvelé leur confiance en l'État français et ont signifié leur volonté d'appartenir à notre nation. Nous ne saurions leur répondre en les considérant comme des citoyens de seconde zone ! Puisque ce budget manque d'ambition, qu'il porte un énième coup de rabot aux services publics ultramarins et ne prend pas suffisamment en compte les spécificités économiques, sanitaires, sociales,

La routine, une année de plus : tout cela parce qu'un énième gouvernement n'a toujours pas compris que, lorsqu'on a entre 23 % et 25 % de chômeurs, tous territoires confondus, et un niveau de revenus inférieur de 10 000 euros à celui du reste du territoire français, il faut sortir de la routine ! Un gouvernement qui n'a toujours pas compris qu'avec des territoires manquant d'infrastructures élémentaires, il faut sortir de la routine Un gouvernement qui n'a toujours pas compris qu'avec une industrie touristique qui pourrait être notre fer de lance, mais dont l'attractivité est en berne, et qui peine à faire face à la concurrence mondiale féroce, il faut sortir de la routine Un gouvernement qui n'a toujours pas compris qu'avec des territoires dans lesquels l'investissement de l'État par habitant est très inférieur à ce qu'il est dans le reste du territoire, il faut sortir de la routine Un gouvernement qui n'a toujours pas compris que, avec des territoires où plus de la moitié de la jeunesse est durablement installée dans le chômage, il faut sortir de la routine qu'avec des territoires, comme la Guadeloupe et la Martinique, où entre 3 000 et 5 000 personnes quittent le pays et, pour l'essentiel, n'y reviennent pas, il faut sortir de la routine

me hurle un énième : « Nous gardons le cap ! » Ce fameux « Nous gardons le cap ! » qui entraîne aujourd'hui des milliers de Français dans la rue. Madame la ministre, nous essaierons de faire. Dans nos pays, nous avons l'habitude de la résignation,

J'ai envie de vous demander, pour parodier une célèbre publicité : Pour toutes ces raisons, madame la ministre, je vous annonce, la mort dans l'âme, que je voterai contre le budget de la mission « Outre-mer

Mais, comme l'ont souligné les rapporteurs, en soustrayant les mesures de périmètre, il apparaît que les crédits de la mission sont en réalité stables, tant en autorisations d'engagement qu'en crédits de paiement. Cela est insuffisant, madame la ministre, pour répondre aux situations difficiles que connaissent nos territoires ultramarins, depuis très longtemps. Une augmentation des crédits aurait été nécessaire pour montrer à nos populations que le Gouvernement avait pris la mesure de leurs difficultés tant structurelles que conjoncturelles. Malheureusement, budget après budget, ministre après ministre, nous sommes obligés de nous battre avec acharnement pour, simplement, conserver l'existant, déjà insuffisant ... L'augmentation du nombre de contribuables à l'impôt sur le revenu par la modification de l'abattement de 30 % et l'augmentation de la taxation sur le rhum, largement infondée, sont symptomatiques des incohérences et des incompréhensions dont fait preuve le Gouvernement en prenant des décisions unilatérales, le plus souvent ministre, lorsque vous évoquez une mesure de santé publique, comprenez notre désarroi dans un contexte où, parallèlement, nous ne savons toujours pas si les taux de sucre dans les denrées alimentaires dans les outre-mer sont bel et bien contrôlés, plus de deux ans après le vote de la loi et la publication, bien tardive, du décret d'application. Comment peut-il y avoir, d'un côté, un empressement à taxer et, de l'autre, un manque de suivi dans l'application d'une loi pourtant fondamentale pour la santé publique ?

Il en a été de même pour arracher des mesures en faveur du logement social et de la rénovation hôtelière. Madame la ministre, j'espère que vous aurez entendu mon message et celui que le Sénat a voulu vous adresser en adoptant ces deux amendements.

Puissions-nous être un jour entendus. Alors les outre-mer ne seront plus considérés comme une charge, mais bien au contraire comme une chance pour la France, un atout supplémentaire pour sa cohésion nationale et son rayonnement international

nous examinons ce matin les crédits de la mission « Outre-mer ». Ce rendez-vous incontournable est l'occasion de nous prononcer sur les orientations politiques et budgétaires pour nos territoires ultramarins. Je tiens avant tout à saluer le travail des rapporteurs, plus particulièrement de mes collègues centristes Mme Dindar, rapporteur pour avis, et M. Laurey, rapporteur spécial. Il est Il est difficile de prendre position sur une mission aussi vaste, avec des domaines divers et des territoires qui ont chacun leurs spécificités.

Cela devrait nous amener à une réflexion sur l'organisation du budget des outre-mer. En effet, cette mission est la seule à vocation géographique. Or nous devrions davantage intégrer les outre-mer dans toutes les composantes du budget. Nous pourrions aussi améliorer la lisibilité de ce budget, pour en avoir une vision plus globale et mieux adaptée à la diversité des territoires. Sur le fond, les défis pour les outre-mer sont nombreux. La situation actuelle à La Réunion est très préoccupante. Les taux de pauvreté et de chômage, bien plus élevés que dans l'Hexagone, ajoutés à la cherté de la vie, ont amplifié et fait prendre une tournure violente au mouvement des « gilets jaunes ». Cette situation met en lumière les difficultés économiques, sanitaires, sociales et sécuritaires auxquelles nombre de territoires ultramarins sont confrontés. Dans ce contexte difficile, ce budget doit avant tout permettre la mise en oeuvre du Livre bleu, fruit des assises de l'outre-mer et remis au Président de la République en juin dernier. Nous en attendons cette année les premières concrétisations. Nous saluons cette initiative, mais nous serons attentifs à leur traduction concrète sur le terrain.

elle s'explique en réalité par des mesures de périmètre qui font évoluer les contours de la mission, ainsi que par trois sources de financement qui existaient déjà, mais dont la nature change. La première de ces sources est la transformation du CICE en exonérations de charges à l'échelle nationale. Les deux autres, ce sont les 170 millions d'euros d'aides fiscales transformées en soutien budgétaire : 100 millions d'euros issus de la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable, 70 millions d'euros de la diminution de l'abattement sur l'impôt sur le revenu applicable dans certains départements et régions d'outre-mer. En définitive, les crédits de la mission « Outre-mer » sont donc stables. La disparition d'aides fiscales a logiquement suscité des inquiétudes chez bon nombre de nos collègues ultramarins. Je crois qu'elle aurait mérité davantage de pédagogie de la part du Gouvernement. Je salue néanmoins, madame la ministre, votre volonté de faire autrement, en changeant le mode d'accompagnement des territoires d'outre-mer. En matière de logement, ainsi que l'a indiqué notre collègue Nuihau Laurey, rapporteur spécial, les moyens budgétaires visant à le favoriser sont stables, mais inférieurs aux besoins. Dans les collectivités du Pacifique, par exemple, les coûts de construction des logements sont très élevés, du fait de l'insularité et de l'éloignement. L'État doit pouvoir apporter un soutien plus actif à ses territoires les plus éloignés. À l'Assemblée nationale, la défiscalisation applicable au secteur du logement social a été étendue aux travaux de rénovation d'immeubles de plus de vingt ans dans certaines zones prioritaires des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. C'est une avancée, mais c'est encore insuffisant. Étant donné les coûts de construction élevés, il faudrait relever le plafond du montant des travaux pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt par logement.

Je tiens à saluer l'implication de l'État, qui a fait en sorte que la consultation se déroule dans les meilleures conditions. Nous avons franchi une étape de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Il faut désormais nous intéresser à son développement économique,

Monsieur le président, mes chers collègues, la trajectoire de politique économique pour les outre-mer que vous nous présentez, madame la ministre, au cours de cette séquence budgétaire, ainsi que les mécanismes qui y président, ont suscité des inquiétudes d'une rare intensité. au cours des nombreuses auditions que j'ai conduites, toutes les remontées de terrain ont convergé pour exprimer de très sérieux doutes sur les choix stratégiques opérés. Au centre de cette politique, c'est la question du développement des outre-mer qui se pose. Ce développement implique une vision de long terme. Or plusieurs points constituent des signaux d'alerte. Le premier concerne la réforme des allégements de charges patronales, un paramètre essentiel pour la compétitivité des économies ultramarines. Si, face à la concurrence régionale et au niveau très bas du coût du travail, cette mesure se justifie, elle ne peut plus se comprendre si l'on se place sur le long terme. De plus, associée à la remise en cause de la baisse des charges sur les salaires d'encadrement et d'expertise, elle enferme les marchés ultramarins, les condamnant à s'inscrire sur des segments de basse et de moyenne gamme. Surtout, cette orientation n'est pas cohérente avec une politique de développement de la formation et d'exhortation des jeunes à participer à la mobilisation économique. Les crédits de l'aide à la formation et à la qualification professionnelles sont, à cet égard, en légère hausse, ce dont il faut se féliciter. Mais, faute de salaires attractifs, trop de jeunes diplômés choisiront de poursuivre leur carrière à l'étranger. Il faut plus globalement prendre garde au nivellement salarial provoqué par une telle politique. Il me semble que le niveau du coût du travail touche à des sujets de fond. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse pour rappeler que, s'agissant de la formation de base, les outre-mer sont pionniers avec un service militaire adapté, le SMA, qui démontre année après année son efficacité.

Fort pertinemment, les travaux du Sénat ont permis de borner la discussion sur l'établissement des seuils d'exonération, qui a été poursuivie durant la navette et à laquelle, madame la ministre, vous vous étiez engagée, l'honnêteté commande de le souligner. Les échanges ont abouti à un relèvement des seuils qui, sans répondre intégralement aux demandes formulées par les socioprofessionnels, constitue une amélioration par rapport au dispositif initial. Je crois pouvoir dire que toutes les collectivités ont exprimé un besoin d'adaptation aux réalités locales, dans un souci d'efficience des dispositifs. Tel a été le cas à Saint-Barthélemy qui a souhaité faire prévaloir la stabilité, surtout dans un contexte économique qui reste, malgré une reconstruction avancée, marqué par l'après-Irma. Saint-Barthélemy n'est pas bénéficiaire du CICE : elle n'était donc pas directement concernée par les enjeux de sa transformation en baisse de charges, et je vous sais gré, madame la ministre, d'avoir entendu cette demande.

Pour 2019, en effet, le budget opère une ponction de sommes disponibles entre les mains des agents économiques pour les centraliser : cela s'appelle une hausse de la fiscalité, qui va modifier les comportements économiques dans un sens restrictif.

Dans ces économies qui peinent, les augmentations fiscales résultant, d'une part, de la réduction de la réfaction de l'impôt sur le revenu des classes moyennes et, d'autre part, de la suppression de la TVA non perçue récupérable, la TVA-NPR, ne pourront avoir qu'un effet déstabilisateur. Avec la réduction de l'abattement de l'impôt sur le revenu, il reste que ce sont 70 millions d'euros dont seront privés des secteurs d'activité tels que les loisirs, les services à la personne, et j'en passe. Dans cette hypothèse, un cercle vicieux, qui pourrait se traduire à terme par une augmentation des dépenses sociales, En outre, bien que n'ayant pas une inclination particulière pour le développement subventionné, il n'en demeure pas moins que la TVA-NPR constitue un élément de la trésorerie des entreprises. Il y a donc fort à parier que celles-ci seront tentées de compenser sa suppression par des augmentations de prix, créant un autre cercle vicieux inflationniste. Il est vrai que les territoires ultramarins se caractérisent par leurs besoins en infrastructures. La progression du fonds exceptionnel d'investissement, dont les crédits s'établissent à 110 millions d'euros, est conforme aux préconisations du Livre bleu outre-mer. Ainsi, à la dépense fiscale faisant appel au libre arbitre des agents économiques, vous préférez la recentralisation des crédits et l'étatisation de la dépense. Le choix a donc été fait de prendre un risque récessif pour améliorer les infrastructures. Là encore, la compensation soulève de nombreuses inquiétudes essentiellement, très prosaïquement d'ailleurs, en raison du traitement administratif des demandes de financement qui seront présentées. Qui va les traiter, à quel rythme et selon quel processus ? Dans Dans tous les cas, entreprises et collectivités auront à remplir des dossiers qui devront ensuite être instruits, cette dernière étape comportant des incertitudes et entraînant des délais d'attente. Madame la ministre, le Gouvernement est-il en mesure de s'engager à des démarches ? L'annualité budgétaire se traduit trop souvent par des crédits non consommés et l'étape administrative ne doit en aucun cas se transformer en une variable de limitation de la consommation. La stabilité du cadre fiscal et économique est l'autre enjeu pour les outre-mer. Chaque gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, se fait fort de présenter sa réforme avant même que les mesures adoptées par ses prédécesseurs n'aient atteint leur rythme de croisière. C'est un incessant qui incessant qui pousse les investisseurs à l'attentisme. Il en va ainsi du CICE, transformé en réduction de cotisations, alors que les entreprises venaient à peine de s'y adapter. Au surplus, cette transformation ne sera pas dénuée de conséquences fiscales. À la différence du CICE, c'est-à-dire un crédit d'impôt assis sur la masse salariale, les baisses de cotisations entraînent une hausse du résultat net et du bénéfice imposable de l'entreprise. Fiscalement, il n'est donc pas certain que les réductions de charges ne soient pas atténuées dans certains cas par des augmentations d'impôts. Par ailleurs, en ce qui concerne les zones franches d'activité nouvelle génération, il conviendra de même d'être attentif aux effets d'éviction qui pourraient être occasionnés par la simplification du dispositif et la suppression des zones géographiques, ainsi qu'aux « trous dans la raquette », comme a pu le redouter un entrepreneur auditionné. Au total, en dépit de toutes les réserves exprimées, je vous fais crédit, madame la ministre, d'avoir pris en compte l'apport du Sénat pour rééquilibrer une approche trop comptable des outre-mer. C'est dans cet esprit constructif que je ne m'opposerai pas à l'adoption de cette mission, espérant qu'elle permettra une coconstruction accrue dans l'unique intérêt des outre-mer. Si, sur un plan purement comptable, notre groupe choisit de ne pas s'opposer à votre budget, reconnaissons ici que, derrière les chiffres, il existe des choix politiques forts et surprenants, pour ne pas dire inquiétants, faits par votre gouvernement. Je peux donc comprendre et partager les inquiétudes qui se sont généralisées en outre-mer. Tout en affirmant votre volonté d'appliquer une politique de différenciation territoriale, madame la ministre, je constate avec une certaine amertume que vous choisissez une direction et un cap diamétralement opposés. opposés. C'est dans les territoires que se prennent les bonnes décisions, c'est dans les territoires que se prennent les décisions les mieux adaptées et les plus efficaces. Alors, pourquoi ne pas laisser et redonner aux territoires les moyens et la liberté d'agir ?

La parole Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la mission « Outre-mer » s'inscrit dans un contexte de maîtrise de la dépense publique. Pour autant, elle n'exclut pas l'ambition d'aider chaque territoire à construire son propre modèle de développement en créant les conditions pour que les initiatives s'expriment et soient soutenues de façon pragmatique, mais durable. Le Livre bleu outre-mer, remis en juin dernier au Président de la République, constitue la feuille de route du Gouvernement pour les prochaines années. Cette mission en est une première traduction financière. C'est pourquoi, à un budget 2018 de transition, succède un budget 2019 de transformation et de responsabilisation. Il s'agit de dépenser mieux pour plus d'efficacité, avec des objectifs prioritaires tels que le développement des infrastructures indispensables au quotidien de la population et au fonctionnement des entreprises créatrices d'emplois et de richesses, mais aussi la réorganisation de l'aide à l'activité économique, la construction et la rénovation de logements et, enfin, la formation des jeunes. Je rappelle que la mission ne couvre qu'un dixième de l'effort financier global de l'État pour les outre-mer. Celui-ci s'élève à plus de 23 milliards d'euros en autorisations d'engagement et à plus de 22 milliards d'euros d'euros en crédits de paiement, soit des hausses respectives de 7,6 % et de 4,6 %. La mission en elle-même, plus de 23 milliards d'euros en autorisations d'engagement et à plus de 22 milliards d'euros

et 0,40 % en 2017, ce qui témoigne de la préservation des crédits spécifiquement affectés aux outre-mer. Les hausses de crédits de la mission 22,5 % en autorisations d'engagement et de 20,52 % en crédits de paiement s'expliquent par des mesures de transfert et de périmètre, conséquences de votre volonté, madame la ministre, de mettre la dépense publique au service du plus grand nombre et de repenser les mécanismes d'accompagnement des économies d'outre-mer. Ces mesures résultent de trois réformes majeures la transformation nationale du CICE en exonérations de charges ciblées sur des secteurs en développement, la suppression de la TVA non perçue récupérable et non perçue récupérable et la diminution du plafond de la réduction d'impôt pour les plus hauts revenus dans les DOM. Ces changements, fussent-ils justifiés par un souci de justice et d'efficience économique, ne se font pas sans appréhension. Ils ont donné lieu à d'intenses débats sur nos travées et sur les bancs de l'Assemblée nationale. Certains craignent que des entreprises soient perdantes, que des territoires ne perdent de l'attractivité, que le pouvoir d'achat ne baisse. promettez de redéployer l'équivalent des euros ainsi obtenus aux outre-mer. Beaucoup voient un changement de paradigme : les outre-mer, dont les handicaps structurels et la légitimité à revendiquer une égalité réelle avec l'Hexagone sont indéniables, s'autofinanceraient dorénavant entre eux, les moins faibles aidant les plus pauvres. Or, vous l'avez dit, madame la ministre, l'État ne se désengage pas. 17 milliards euros de crédits aux outre-mer, bien que la fiscalité n'y rapporte que 4 milliards d'euros. J'ajoute que cet effort est largement fondé, ne serait-ce qu'en raison

Nous attendons que la réduction des dépenses fiscales et sociales se traduise bien en dépenses budgétaires et pilotables. Les économies issues de la suppression de la TVA-NPR alimenteront le programme 138 de la mission pour améliorer l'accès au financement des entreprises. J'espère aussi que le fonds exceptionnel d'investissement du programme 123 ainsi abondé sera utilisé et ne perdra pas de sa substance au fil des années. Je l'attends d'autant plus qu'une partie de ce fonds doit être consacrée à la construction d'établissements scolaires en Guyane et à Mayotte. J'aurai l'occasion d'y revenir lors de l'examen de la mission « Enseignement scolaire ». Le nouveau dispositif de zones franches, simplifié et ciblé sur des secteurs d'activités soumis à la concurrence, mais essentiels par leur capacité à créer activité et emplois, contribuera à la revitalisation des économies ultramarines. Tout en restant ferme dans vos convictions, vous avez su écouter nos inquiétudes et apporter des ajustements, madame la ministre. Vous avez modifié les paramètres des nouvelles exonérations de charges pour les entreprises, afin d'atténuer le phénomène de trappe à bas salaires. Vous avez élargi les secteurs éligibles. Vous avez tenu compte des particularités de la Guyane, notamment. J'insiste, nos territoires d'outre-mer restent fragiles. Cette fragilité recouvre des difficultés parfois semblables, parfois de nature très différente. Promouvoir un développement endogène est vertueux, mais veillons à ce que des outils mal ajustés ou mal des outils mal ajustés ou mal compris ne nous entraînent pas dans une logique de mal-développement endogène. La crise qui a bloqué Mayotte plusieurs mois durant a révélé l'importance du contexte régional dans la conduite des politiques publiques locales. Mayotte, qui fait face à une très forte immigration, a montré qu'elle manquait cruellement de sécurité, de logements, d'écoles, de routes et d'un aéroport adapté- j'insiste sur ce dernier point. Dès lors, attirer les compétences et les y maintenir ? Très récemment, les Réunionnais ont montré leur profond mal-être. Madame la ministre, vous êtes allée à leur rencontre et avez annoncé des mesures, dont plusieurs sont d'ailleurs déjà inscrites dans le budget de l'État. Vous avez ainsi annoncé la création d'une zone franche globale à 7 % à La Réunion.

Les besoins en logements sont considérables. Il faudrait en construire 50 000 en Guadeloupe d'ici à 2030, plus de 4 000 par an pendant vingt ans en Guyane. À Mayotte, seuls 570 logements locatifs sociaux et très sociaux ont été financés entre 2015 et 2017. Les déplacements ultramarins du Président de la République et de nombreux ministres témoignent de l'intérêt de la Nation pour les outre-mer. À la suite de ce premier budget de transformation, les budgets qui lui succéderont continueront d'y apporter, je l'espère-

Notre combat, jusqu'ici, a été de tenter un rattrapage à tous les niveaux des départements d'outre-mer vers la métropole. Tout s'est passé comme si, dans l'Hexagone, cette volonté procédait d'un souhait utopique.

madame la ministre, c'est à regret que je relaie ici les inquiétudes suscitées par votre budget, tant il est crucial pour nos collectivités de sortir de l'incompréhension qui mène au mal-développement. Après plusieurs longs mois d'assises des outre-mer, la déception est d'autant plus grande que les attentes se sont exprimées directement à partir des territoires, qui savent assurément ce qui est bon pour eux. Mes collègues ayant déjà évoqué avec pertinence les aspects purement budgétaires, je veux, dans le temps qui m'est imparti, me concentrer sur l'état d'esprit qui préside à la politique économique de votre gouvernement, dont nous examinons la traduction chiffrée aujourd'hui.

Localement, la redéfinition des seuils d'exonération, dont les crédits de compensation nous sont présentés, laisse le sentiment amer d'un gouvernement sourd à la vision des socioprofessionnels ultramarins. Pis, le recentrage de nos économies sur les bas salaires risque de pénaliser plus encore une jeunesse déjà fragile et en mal de débouchés. L'augmentation des crédits de cette mission résulte donc essentiellement d'un jeu d'écritures, inscrivant ici des crédits qui auraient pu l'être ailleurs, dans d'autres missions. En outre, le « recyclage » mentionné par le président Magras « rebudgétisation » dénoncée il y a quelques jours par le sénateur Lurel inaugurent une rupture brutale de la solidarité nationale à l'endroit des outre-mer. Dès lors se pose une question de fond, qui va bien au-delà de la simple annualité budgétaire du maintien d'un ministère spécifique des outre-mer. À mon sens, ce ministère est certes un gage de sanctuarisation budgétaire, mais c'est aussi un « plafond de verre », qui nous enferme dans un entre-soi, qui ne parle de nous-mêmes qu'à nous-mêmes.

Ainsi, au fil des années, à périmètre constant, cette enveloppe stagne en réalité autour de 2,5 milliards d'euros alors que, dans le même temps, la question du développement endogène de nos différents territoires se pose avec beaucoup plus d'acuité. Je sais combien la tâche est madame la ministre, et que vous vous investissez sans relâche. Pour autant, je ne peux pas approuver les orientations de ce budget ni m'empêcher de penser, en conscience, est peut-être temps d'emprunter d'autres voies, notamment institutionnelles. Je souhaite conclure par ces mots de Frantz Fanon : « La politisation des masses se propose non d'infantiliser les masses mais de les rendre adultes. » La parole

La parole

Pour autant, il faut aussi de la lucidité, pour reprendre une expression présidentielle, mais cette fois-ci de notre président, Gérard Larcher. À un moment donné, si le bateau gouvernemental ne suit pas la boussole, qui est celle du CROSS Étel et, en l'occurrence, la boussole parlementaire qui donne un certain nombre de signaux, il s'échoue sur les rochers ou sur les coraux.

Je suis inquiet pour mon territoire, comme je le suis pour le reste des territoires d'outre-mer, compte tenu de la méthode employée et des crédits engagés. J'espère, madame la ministre, que vous pourrez apporter un certain nombre de réponses de nature à rassurer mes collègues du groupe du RDSE. Aujourd'hui, nous sommes réservés sur cette mission parce que, comme l'a rappelé Guillaume Arnell, nous avons ces inquiétudes.

vous le savez, je reviens tout juste d'un déplacement à La Réunion. Je suis allé au contact de la population, parce que la seule méthode qui ait du sens pour moi, c'est l'écoute et le dialogue avec nos concitoyens.

Paris, aujourd'hui, notre modèle de vivre-ensemble, qui a tant fait notre fierté, est mis à mal. C'est dans ces moments que le mot « gouverner » » doit prendre tout son sens : gouverner, ce n'est pas imposer d'en haut des choix déconnectés de la réalité du terrain ; c'est toujours agir en responsabilité, guidé par l'intérêt général, pour que chaque citoyen trouve sa place dans la société.

L'État a pris des engagements forts et je rendrai compte de leur mise en oeuvre à La Réunion et dans tous les territoires, tout comme je veillerai d'ailleurs à ce que chacun joue le jeu républicain. Cette responsabilité et cette transparence sont à la base de mon action. Vous le savez tous, depuis dix-huit mois, je travaille pour transformer nos territoires dans la dignité, le respect et l'unité, pour des outre-mer pleinement inscrits au coeur de la République. Le projet de budget que je vous présente découle bien sûr de choix politiques majeurs et de convictions fortes. Ce choix de la transformation, c'est le refus du conservatisme, c'est la volonté d'accompagner les territoires vers un développement qu'ils auront eux-mêmes défini. C'est le propre de la démocratie participative et ce besoin s'est clairement exprimé sur le terrain, ces jours derniers. C'était l'intérêt premier des assises des outre-mer : l'expression directe de milliers de citoyens, d'entrepreneurs, de porteurs de projets, qui nous disent à quel point l'État est attendu ! Ce n'est pas toujours plus d'État, mais mieux d'État Les exaspérations, les inégalités, les injustices exprimées, je les comprends comme une incitation à aller plus loin et à poursuivre dans la voie de la transformation.

l'emploi. Oui, l'emploi est une priorité parce que, sans activité, sans travail, sans fierté, un territoire, quel qu'il soit d'ailleurs, n'est qu'un navire à la dérive avec un équipage totalement perdu, et souvent en colère. Il y a le pouvoir d'achat,

Face à ces aspirations, je ne promets pas une égalité réelle ni une convergence des niveaux de vie vers une moyenne nationale, dont tout le monde sait que celle-ci recouvre Ce n'est pas ma vision des choses, vous le savez. Chaque territoire ultramarin doit trouver son propre modèle de développement. Et comme je le rappelais à La Réunion, l'État ne fera pas seul. Il n'est pas, tant s'en faut, le seul à détenir les réponses aux défis qui sont devant nous. Pour permettre aux territoires d'enclencher cette dynamique de progrès économique, le présent projet de budget nous donne les moyens d'agir sur l'investissement public et d'appuyer les entreprises. l'investissement public, les crédits du fonds exceptionnel d'investissement sont portés de 40 millions d'euros à 110 millions d'euros par an. Ce niveau d'engagement sera maintenu tout au long du quinquennat. Sur cinq ans, ce sont donc 500 millions

Ces contrats de convergence vont s'accompagner du mot « transformation ». Ils seront signés dans les prochaines semaines et scelleront les engagements de l'État et des collectivités jusqu'en 2022. Les outre-mer sont en avance sur l'Hexagone : quatre ans, l'effort de l'ensemble des périmètres ministériels va s'élever à 2 milliards d'euros. Pour ce qui est du ministère des outre-mer, nous allons y consacrer 179 millions d'euros en 2019, soit 15 % de plus que l'an passé. L'investissement public, c'est également la construction et la rénovation de logements. Vous avez raison, mesdames, messieurs les sénateurs, il s'agit d'une préoccupation essentielle dans les territoires d'outre-mer. La ligne budgétaire unique

j'ai eu l'occasion de réaffirmer les engagements pris en matière d'accession à la propriété et d'aide à la rénovation de l'habitat privé : traitement de l'ensemble des dossiers actuellement bloqués,

Je crois que la réponse ne peut pas être que sociale, comme vous le savez tous ici. D'ailleurs, le présent projet de loi de finances comporte de nombreuses mesures fiscales favorables à la construction de logements : prolongation de la défiscalisation, amélioration de la chronicité du versement du crédit d'impôt, mais aussi augmentation des quotas de allongement des délais de mise en location ou encore extension de la défiscalisation dans les collectivités d'outre-mer pour la réhabilitation du parc social existant. Accroître l'investissement public est fondamental pour répondre aux besoins du quotidien des Ultramarins.

Depuis décembre 2017, le Gouvernement a proposé de faire évoluer les aides pour l'emploi et l'activité économique outre-mer. Vous le savez, un travail énorme a été mené en ce sens. L'objectif était bien de définir une politique de développement économique volontaire, pilotée et cohérente et d'inscrire les dispositifs d'accompagnement dans le temps long. Oui, certains outils disparaissent, parce qu'ils ne sont pas assez lisibles, parce que l'on ne savait pas, au final, où allaient véritablement les financements, parce qu'ils ne servaient qu'à quelques-uns,

Notre objectif n'a pas varié sur la question de l'écosystème d'accompagnement des entreprises : ce système doit être pérenne et ciblé, afin de faire des outre-mer des territoires de conquête économique. Si nous voulons l'excellence, nous devons être à la hauteur ! La transformation du CICE en allégement renforcé de charges sociales a entraîné un bouleversement des exonérations spécifiques aux outre-mer. Dans ce contexte, notre volonté a été d'assumer une politique de l'emploi,

Nous avons mené un travail approfondi avec les administrations et les professionnels. Le Gouvernement a réalisé un effort supplémentaire de l'ordre de 130 millions d'euros, afin d'abaisser le coût du travail en outre-mer, tout en conservant l'objectif de mener une politique volontariste pour l'emploi et contre et contre le travail illégal. Les conséquences budgétaires sont tirées sur la mission « Outre-mer ». Tel est le sens des amendements qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale, avec 30 millions d'euros

qu'il nous fallait encore travailler, et jusqu'au dernier jour, avec l'ensemble du monde économique et coller à la réalité des besoins des territoires. C'est ce que nous avons fait à ce stade. Je précise que la modification des circuits de financement des exonérations de charges a entraîné une mesure de périmètre, faisant entrer 300 millions d'euros dans notre budget. Il s'agit d'une mesure purement technique. Vous connaissez ma volonté de transparence

Pour améliorer le financement de l'économie, la mission « Outre-mer » sera enrichie de nouveaux outils nécessaires au démarrage des projets. C'est l'objet de la nouvelle action n° 04, qui figure désormais au sein du programme 138. Avec la réforme des dispositifs zonés et la prolongation de la défiscalisation, nous allons construire un ensemble cohérent et efficace. mesurer les conséquences. S'y ajoute le renforcement des moyens dédiés au financement des investissements structurants, qui bénéficient directement à l'activité des entreprises, puisque, vous le savez, construire des écoles

! Comment faire mieux pour permettre l'excellence dans les territoires d'outre-mer ? Démontrons tous ensemble que nous sommes capables de relever le défi qui nous est posé. Mesdames, messieurs les sénateurs, conformément aux orientations du Livre bleu, ce projet de budget propose de transformer nos territoires pour les rendre plus attractifs, plus agréables à vivre, pour en faire des terres d'excellence et de rayonnement, car, oui, nous sommes des richesses. Être une richesse,

ne pourra être opérationnelle que si l'ensemble de la classe politique des territoires d'outre-mer, mais aussi de nos acteurs sur le terrain travaillent à une logique collective de construction. les Réunionnaises et les Réunionnais nous l'ont montré, les Ultramarins sont exigeants. Et ils ont raison de l'être ! Je le suis moi-même.

Nous devons être à la hauteur des valeurs qui sont au fondement de notre vivre-ensemble : la fierté, l'unité, la dignité et la fraternité. Ces valeurs sont le socle de l'esprit républicain, l'essence même de la France des outre-mer. Nous allons

maintien des spécificités de la Guyane, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Nous allons consentir un effort supplémentaire de près de 100 millions d'euros sur le budget de la Nation.

peuvent exister entre nos territoires, nous sommes capables d'aller au-delà de nos divergences et de trouver un terrain d'entente. J'ai eu à défendre

J'avoue que nous sommes assez surpris, outre-mer, du peu d'importance accordée par le Gouvernement à ce qui nous paraissait un concept novateur.

et de mobilisation à destination des populations, des entreprises, des collectivités locales et de toutes les forces de secours, à l'instar de la sécurité civile, afin de garantir des capacités d'intervention rapide et efficace sur les territoires. Il s'agit, par ce plan, d'une part, de renforcer l'acquisition de moyens

dans les territoires, une « semaine des risques naturels majeurs » sur le modèle de REPLIK ou de SISMIK, avec des outils, des dispositifs et des messages spécifiques à chaque territoire, tels que la prévention en milieu scolaire ou des exercices de simulation d'aléas. Des moyens supplémentaires aux différents dispositifs existants sont donc nécessaires pour anticiper et prévenir les dégâts et les pertes humaines évitables. Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence

manière récurrente, en particulier pour ce qui concerne le transport aérien. Il y a là des améliorations à

un tiens vaut mieux que deux tu l'auras ! Les risques majeurs, c'est tous les jours ! Ce sont des communes qui sont inondées, des personnes qui disparaissent, des travaux importants qu'il faut réaliser dans l'urgence, des moyens dont il faut doter les services de sécurité civile, qui se portent au-devant des populations et se

largement impliqués dans la COP21. Je travaille sur ces sujets depuis de nombreuses années. J'ai répété à plusieurs reprises que le milieu insulaire était la première victime

Ultramarins, qui sont obligés de rechercher en permanence des solutions palliatives. Cette situation, indigne pour une nation comme la nôtre, requiert de la part de la solidarité nationale un engagement massif et urgent pour doter l'ensemble des territoires d'infrastructures adaptées en matière d'assainissement et de distribution d'eau potable.

de la santé, l'Agence française de développement, la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française pour la biodiversité, à accompagner par contractualisation, sur une durée de cinq ans, les collectivités locales compétentes

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à mettre en place un fonds de 10 millions d'euros, en soutien aux services publics des secteurs du sanitaire, du social, de la culture et de la jeunesse. L'action n° 04 destinée à ces domaines n'a bénéficié que d'une augmentation factice de 0,51 %. Vous conviendrez, mes chers collègues, que cette hausse est bien insuffisante pour améliorer de manière réelle les conditions de vie de nos concitoyens ultramarins. Alors que les outre-mer souffrent d'une véritable carence en termes d'investissements et de structures sanitaires, sociales et de loisirs, nous ne pouvons laisser se créer de tels écarts avec la France hexagonale. Nous proposons donc de financer une telle action par la ponction de 10 millions d'euros de l'action n° 09 du programme « Conditions de vie outre-mer », qui ne sert qu'à payer des intérêts bancaires. Les dotations des collectivités publiques étant en baisse et le budget en faveur des services publics stagnant dans ce projet de loi de finances pour 2019, il nous semble plus judicieux d'injecter les financements étatiques dans des actions pouvant impacter positivement le quotidien des Ultramarins. Un tel geste viendrait contrebalancer un budget fortement tourné vers l'investissement afin de redynamiser économiquement ces territoires, où le chômage est élevé et l'emploi précaire. Le problème de la pauvreté ne peut être simplement résolu résolu en donnant une activité professionnelle à tous. D'autres paramètres sont également à prendre en compte, et c'est là le sens de cet amendement. Un soutien accru à l'action n° 04 du programme « Conditions de vie outre-mer » pourrait se révéler salutaire pour des territoires dont les habitants souffrent au quotidien des manques sanitaires et sociaux, mais aussi de l'absence d'infrastructures éducatives, sportives et culturelles. Nulle part sur le territoire de la République l'exécutif ne devrait abandonner ses administrés sujets aux inégalités sociales. Mme Catherine Conconne. Madame la ministre, tout à l'heure, vous avez fait appel aux élus locaux, et moi je partage cette façon de voir. Je ne crois pas en la tutelle bienfaitrice d'une mère patrie qui ferait tout pour nous à notre place et en nous remplaçant. Je crois dans cette main qui cette main qui n'écrase pas, en un cheminement, pacifique, serein, entre les populations de ladite outre-mer et l'État central. Alors, madame la ministre, avec cet amendement, je vous prends au mot. Le poète a dit : « Gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur. » Nos pays, la Guadeloupe et la Martinique, vivent un vrai drame : le dépeuplement.

Vous imaginez l'impact sur la démographie : la population vieillit, puisque cette population jeune qui s'en va, c'est celle qui assure, en quelque sorte, par sa fertilité, le repeuplement.

Nous avons besoin de vous, madame la ministre. Le travail a été mené en amont et les populations martiniquaises ont oeuvré en faveur de ces propositions.

Les retards de paiement dans les départements et régions d'outre-mer restent courants. Par exemple, en 2016, 40 % des entreprises ultramarines subissaient un tel retard. Elles étaient par ailleurs 45 % à régler leurs fournisseurs au-delà de 60 jours. Les retards de paiement ont donc un impact important sur la trésorerie des entreprises. Celles-ci peuvent être incitées à reporter le règlement de leurs factures. Les délais de paiement des entreprises domiennes sont ainsi supérieurs à la moyenne nationale 63 jours d'achat contre 51 jours pour les délais fournisseurs, et 54 jours de chiffre d'affaires contre 44 jours pour les délais clients. Les délais fournisseurs restent eux aussi supérieurs à la valeur de 60 jours d'achat prise comme estimation de la limite légale de 60 jours de règlement introduite par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. De la même manière, le délai légal de paiement pour les collectivités territoriales est de 30 jours ; dans les faits, il est en moyenne de 28 jours en France hexagonale. Il atteint toutefois 74 jours en Guadeloupe, 115 jours en Martinique, 86 jours en Guyane, 45 jours à La Réunion et 57 jours à Mayotte. Dans des territoires où les marchés sont étroits et au sein desquels le poids de la commande publique dans l'économie est prépondérant, il est délicat pour les entreprises de demander aux services de l'État des mandatements d'office. Il est par conséquent urgent que l'État dresse un bilan clair de l'état des retards de paiement dans ces territoires et qu'il établisse un ordre de priorité des dépenses à payer. À plus long terme, les dispositions prévues pour éviter les retards de paiement n'ayant pas permis d'éviter les dérives actuelles, il conviendrait d'engager une réflexion plus générale sur une éventuelle refonte les concernant.